La séance est reprise nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 dont le Sénat et saisi en application. L'article 47, un alinéa de la Constitution dans l'édition des articles nous sommes parvenus à l'article 19. Mais avant que nous entamions édition des Arctic. La parole est donnée à madame Nadia le groupe pour une mise au point, au sujet d'un vote. Oui madame la présidente, je souhaite procéder à de rectification de vote lors du scrutin, numéro 203 du 7 mars. Mon collègue Jean Marie la Rimbert souhaitait s'abstenir et lors du scrutin, numéro 247 du 9 mars, ma collègue Christine Herzog souhaitée également. Sonia je vous remercie.

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les cotisations sont au coeur du problème de financement du système de retraite. Une des raisons essentielles. Qui explique le manque de recettes. C'est la suppression de l'emploi public. Les atteintes que ceci implique à l'emploi tit territorial et hospitalier. Qui généreront d'ailleurs autant de déficit. La baisse des rémunérations de l'emploi public sera diminué aussi en proportion des rémunérations totales. Par conséquent ce sont les recours massif aux contractuels.

Le gouvernement en est pleinement responsable. C'est sa feuille de route austéritaire transmise à Bruxelles dans le cadre du programme de stabilité qui acte le désengagement de l'emploi public et donc le déficit de retraite qu'il se propose de réformer, c'est bien la logique du pompier pyromane, que le gouvernement applique à ce bien commun ce bien précieux qu'est notre système de retraite. À contrario, notre groupe est porteur de propositions. Que je rappellerai ici rapidement. L'augmentation des cotisations qui aurait pesé un vrai segments sur les bords revue moins sur les bas revenus. de rémunération des accessoires de rémunération que sont la participation l'intéressement. L'augmentation de la CSG sur le capital. L'augmentation de la contribution sociale de soleil solidarité etc la liste serait bien entendu plus longue mais pour se convaincre des possibilités de financer autrement. Il suffit de se rappeler. Le titre D'un grand quotidien du soir dans son édition d'hier. Qui nous ne pourrait nous donner quelque inspiration sur la mise à contribution. Des revenus par exemple du CAC 40. Merci de votre attention. Merci madame Le Houerou. Merci madame la présidente. comme les allocations du minimum vieillesse, aux personnes âgées pour tous les régimes de retraite qui en assure le service selon l'adresse en 2019 75 % des allocataires du minimum vieillesse vivent plus souvent seuls, 54% des allocataires sont des femmes, l'âge moyen des allocataires et de 74 ans. Le fonds de solidarité vieillesse finance aussi les dépenses liées à la prise en charge sur des bases forfaitaires de cotisations de retraite au titre de la validation des périodes non travaillées en cas de chômage, le recul de l'âge de 62 à 64 ans creusera davantage les inégalités et allongera le sas de précarité entre emploi et retraite. L'économiste Michaël Zemmour qui nous a beaucoup éclairé pour comprendre les effets de votre réforme. Je le salue. Il nous explique que pour les ouvriers et plus encore les ouvrières, l'allongement du sas de précarité entre emploi et retraite. Elle, elle fait le plus important de la réforme. En 2019, à 61 ans le taux d'emploi des ouvriers et des ouvrières et de seulement 28%, tandis que le taux des ouvriers et des ouvrières ni en emploi, ni en retraite est de 35% selon l'Insee, en 2017, la réforme de 2010, traduite par une hausse de 14. Du taux d'emploi à 60 ans de 13 points du taux de chômage est de 7. Pour l'invalidité et la maladie. Par conséquent, le projet de loi risque d'augmenter pour le FSV. Le fonds de solidarité vieillesse, les dépenses liées à la prise en charge sur des bases forfaitaires de cotisations retraite au titre de la validation des périodes non travaillées en quatre chauvin de chômage ou inactivité globalement vaudrait forme et injuste et injustifiée. Elle doit être retirée.

Merci. Monsieur Chantrel. Merci. Madame le héros.

Merci madame la présidente. Moi je vais faire court Donc c'est ah oui quand même. Article 19, donc c'est effectivement. Une suppression de cet article donc cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicain vise à rejeter la confirmation des prévisions. Des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires F. S. V. tels que le gouvernement l'prévu dans cet article, merci. Merci madame la présidente, chers collègues. Au-delà des projections de de de masse salariale d'inflation. Très faible par rapport à ce que nous disent certains économistes reconnus hein certains qui avancent même qu'on va rentrer dans une période de stagflation de de de de composés d'inflation et de décroissance. Par rapport à l'aune nomme et également qui diminue à à euros constants. C'est-à-dire corrigés de de l'inflation. Le le le paragraphe de de de cet article 19. Elle dit que et je le cite mot pour mot la trajectoire financière traduit la normalisation progressive de la situation sanitaire. Ah très bien. Je pose la question au au ministre. C'est quoi la normalisation sanitaire en matière de sanitaire et de systèmes de santé. Est-ce que vous êtes allés le le dire et l'expliquer sur le terrain au personnel des hôpitaux, des Ehpads, des services d'accompagnement à domicile des services de des infirmiers à domicile. Des personnels des secteurs psychiatriques qui sont en grande difficulté et qui vivent leur situation professionnelle. Comme un abandon de l'État. Voilà allez allez-y, allez leur parler sur le terrain. Vos projections ne sont pas à la hauteur des besoins de financement d'un projet national de santé reconsidérer et conforter. C'est la Razom pour laquelle avec cet amendement. 1300. Nous demandons la la suppression de l'article 19.

Je voudrais simplement noter que. Cet article prévoit une diminution du. Du du Fonds de solidarité vieillesse, alors même que les besoins. Sont importants et et sont devant nous et alors même que pour permettre de à nos personnes personnes âgées de vivre dignement. Il serait souhaitable de revaloriser cette. Cette allocation de de solidarité. C'est une raison supplémentaire pour. pour. Considérer que cette loi est une mauvaise loi sur cet aspect-là en particulier. Et même si elle concerne principalement la la réforme des des des retraites est une réforme qui est vous le savez n'est pas du tout. Acceptée par nos concitoyens à travers les manifestations qu'il a eu au cours de ces derniers

elle ne prend pas en compte les les attentes de nos concitoyens. Et et au surplus, il s'agit d'une sorte de mépris à la fois de nos concitoyens qui ne sont pas entendus, mais également de notre assemblée puisque les différends ont renforcé ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé mais qui est ici aujourd'hui dans le cadre de cette réforme un parlementarisme. Merci. Merci monsieur Tissot. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Mon amendement propose la suppression de cet article 19 qui fixe la prévision de charges de fonds de solidarité vieillesse ce fonds a pour mission de financer divers avantages vieillesse à caractère non contributif qui relèvent de la solidarité nationale. La prévision affichée à cet article 19 ne nous semble pas à la hauteur des besoins aussi faute de pouvoir l'abonder puisque seul le gouvernement a le droit de créer des dépenses dans nos textes budgétaires. Nous voulions ouvrir le débat avec cet amendement de suppression au moment où nous avons déposé nos amendements. Nous ne savions pas encore avec quel mépris le gouvernement les traiter l'opposition sénatoriale et que de débat il n'y en aurait pas. Un maire de mon département consternée par l'absence de réponse de la majorité sénatoriale et du gouvernement dès le début de nos débats m'a suggéré de rester silencieux pendant les deux minutes de mon temps de parole. Cela aurait pu être tenté, ne serait-ce que pour voir si nos collègues de droite se sera aperçue tant ils ont voulu se faire sourd à nos propositions et à nos arguments. Depuis la semaine dernière. Mais avec mes collègues de gauche j'ai préféré continuer à me faire le porte-, parole de nos concitoyens. Ceux-ci sont nombreux à nous écrire chaque jour depuis 2 semaines pour nous demander de vous faire entendre la réalité de ce qu'ils vivent pour essayer de vous faire comprendre que le sacrifice que vous leur demandez ces deux ans de leur vie n'est pas possible à consentir. Hé bien qu'il soit des millions de Français à s'exprimer par tous les moyens à leur disposition compte cette réforme, les sondages d'opinion les raisons socio-les interpellations de leurs élus et bien sûr ces si grandes manifestations. Il ne se. même repris pardon ce même mépris avec lequel le président de la République traite les syndicats qui présente pourtant un front unique historique ce mépris ne fera qu'alimenter la colère de nos concitoyens et conforter leur détermination à mener la bataille jusqu'au bout contre cette réforme et pour paraphraser la chanson entendez le cri sourd du pays qu'on aliène retirez votre projet. Merci. Le 40 64 de madame Assassi. Monsieur. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, puisque vous avez de toute façon acté que nos amendements ne méritait pas d'être mise au vote. Je vais profiter de ma prise de parole pour dénoncer un aspect brutale, inutile de votre réforme. En effet, sur bien des points, notamment en poursuivant la casse des régimes pionnier attachés à des professions dites pénibles, vous vous attaquez notamment aux industries électriques et glacière hein tels qu'EDF à la Régie autonome des transports parisiens, les clercs et employés de notaire, la Banque de France. Les membres du CESE. Vous avez préféré protéger les intérêts des plus privilégiés. Plutôt que de vous attaquer justement à leurs intérêts en dégradant les régimes dits spéciaux, ce que vous faites avec la suppression de ces régimes pionnier est tout simplement insupportable et injuste d'où notre amendement de suppression de je vous remercie. Merci madame Vogel pour le 32 12 à Bruxelles. Retenu par la réunion de la direction du Parti Vert européen dont je suis la coprésidente. Et je sais pas pourquoi ça vous énerve et. Ça m'a donné l'occasion de parler à mes collègues européens de ce qui se passe évidemment en France et je voulais vous dire le quoi qu'on pense des différents systèmes au niveau européen et quelle que soit la position. Les uns et les autres et sur l'âge légal de départ à la retraite en France, en Espagne, en Allemagne, au Danemark ou ailleurs. Chacun et chacune et scandalisés par l'étendue de la violation du débat démocratique en France. Si, manifestations. c'est un fait si manifestations historiques, 90% des actifs, opposé à la retraite à 64 ans et votre seule réponse, c'est le mépris envers l'opposition sénatoriale le mépris du président de la République envers les syndicats. Le mépris envers les salariés et les Français. Nous allons nous retrouver à voter dans cette chambre après un débat hein sincère des abus de procédure sans que l'Assemblée nationale ne se soit prononcée, sans que le président de la République accepte de parler avec l'Dicale avec des millions de personnes descendues dans la rue prêt à parier que personne dans cette chambre très certainement ne va être directement touchés par cette réforme. Avant de conclure, j'aimerais vous demander, malgré tout, et même si. vous ne partagez pas toujours toutes nos idées doute sur tous les bancs d'applaudir en son absence, notre collègue Raymonde Poncet Monge. Pour la conviction l'esprit et les tripes qu'elle a mis dans cette bataille. Je vous remercie. Et d'applaudir aussi ses équipes en général et les nôtres qui pendant des jours et des nuits ont été mobilisés pour ce à quoi elle croit profondément. Je vous remercie. Merci madame la présidente, messieurs les Ministres, chers collègues, la commission en fait se félicite du retour à l'équilibre rapide de du FSV, qui sera à 2 de 8 milliards d'euros d'ici 2026. Et je pense qu'on doit se poser la question d'une réaffectation en fait d'une part de la CSG soit au régime au régime général soit à la cadette. Donc c'est une réflexion que je pose en tout cas, en tout état de cause, la commission a émis un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements de suppression. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente madame la rapporteur, a dit l'essentiel. Je partage et son avis et selon son sentiment sur les réflexions à avoir, par ailleurs, il s'agit d'un article obligatoire dans le cadre de la présentation d'un PLFSS qui interdit d'une certaine manière toute suppression s'sophro rendent le texte absolument impossible à adopter. Merci. Nous passons l'article 20. Les demandes de parole Me Poncet Monge. Madame, Lubat. Merci madame la présidente. Moi je voulais juste au travers de de cet article rappeler que au final. Avec les. Comment dire. Les petites douceurs que le gouvernement aura accepté à la demande. De la majorité du Sénat pour adoucir. Ce projet de loi pour le faire paraître un tout petit peu moins brutal. Ça arrange bien le gouvernement d'un côté s'arrange bien aussi. La majorité sénatoriale bien au final, nous ne savons plus. Ce que va coûter ou rapporter bien que le terme ne me plaisent pas du tout cette réforme elle était faites au départ. Pour économiser 18 milliards d'euros. Je serais bien curieuse de savoir et nous serons bien curieux de savoir d'ici 2 ans, ou trois. Lorsque les chiffres sortiront ce que ça aura clairement à mener, moi je vous le dis. Je pense que cette réforme sera une réforme pour rien au niveau des finances publiques mais coûtera très cher à tous les salariés qui seront concernés. Merci madame la présidente, mes chers collègues. Je voudrais pour ma part, revenir sur le passage. Certes un peu houleux du président de la République récemment au Salon de l'agriculture. Il a pris l'exemple des agriculteurs pour illustrer sa pensée, sa vision du travail et au fond le sens de sa réforme des retraites. Je cite le président. Quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche où il peut se reposer, ils trouvent ça juste. Il aurait pu prendre le président de la République. L'exemple des mineurs de charbon du 19ème siècle pour justifier les régressions de sa réforme en matière de pénibilité ou encore le travail des enfants, c'est au siècle dernier pour présenter l'allongement de la durée de cotisation. Oui, les agriculteurs français ont du mérite et si leur situation vous préoccuper vraiment vous n'auriez pas attendu une proposition de loi des communistes pour revaloriser leurs pensions et à cet égard je veux rendre un hommage particulier à mon collègue André Chassaigne à l'Assemblée nationale pour le travail. pour le travail remarquable qu'il a su mener sur le sujet au fond quel est le sens des mots du président. Il y a des contraintes liées à la profession qui sont indéniables, mais si les agriculteurs travaillent autant sans trêve et si longtemps c'est d'abord parce qu'ils sont mal trop mal rémunérés. Ils sont mal rémunérés pour la même raison que vous faites cette réforme des retraites parce que vous avez choisi votre camp, celui des grands groupes, celui des profits et c'est valable autant pour les. Pétrolier que pour les. Géants de l'agroalimentaire. Alors si vous respectez réellement le travail des agriculteurs indispensable pour notre autonomie alimentaire, ce n'est pas en vous attaquant au régime de retraite de nos concitoyens que vous résoudrait le problème mais bien agissant pour leur assurer une rémunération juste et digne à la hauteur de leurs efforts. Merci beaucoup madame la présidente. Nous arrivons à l'article 20 et cet article il montre hein. Et bien que nous sommes sur la voie de la consolidation de nos régimes de retraite et ça méritait d'être dit. Alors en 2000 en 2023. On le voit, cette réforme elle aussi sociale parce que les mesures d'accompagnement. Elles entrent en vigueur dès le 1er septembre. Ce qui fait que d'ailleurs nous allons dégradé de 300 millions d'euros en 2023. La copie budgétaire mais derrière, hé bien nous allons préserver notre système à l'horizon 2030 puisque dès 2024, dès 2025, on le voit, hé bien le déficit est atténuée et cela, je vais vous dire au au moment où les uns et les autres vous avez rendu hommage à des collègues, hé bien moi je veux rendre hommage aussi à de nombreux collègues qui ici n'ont pas forcément pris la parole. Une heure par jour mais qui mais qui, par leur présence par leur assiduité par le travail en commission hé bien ont voulu apporter leur Pierre à l'édifice de ce sauvetage du système des retraites parce que c'est grâce à eux. Aussi dans quelques minutes, je l'espère, dans quelques heures après peut être d'ultimes. Procédure qui peut être seront utilisées. Eh bien nous permettront de regarder. Nos enfants et nos petits-enfants fassent parce que nous savons que nous aurons agit pour les prochaines années et que c'était indispensable. Alors c'est vrai qu'il est plus facile parfois de tenir le beau rôle mais nous tenons le rôle qui est le nôtre avec fierté et alors que la conviction d'avoir fait le travail qu'il était nécessaire, je vous remercie. Le 394, madame Ferré. Le 546 Monsieur Gillet. Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Article 18, atchik 19. Article 20. Faut-il le rappeler pour cet article qui rajoute 400 millions d'euros mais essentiellement lié à la robe. L'arrestation du minimum contributif. Ah la la revalorisation accordée pour rattraper l'inflation. Cet article en fait il illustre aussi tout le système complexe que l'on essaye de mettre en place en terme de filet de sécurité, de politique de solidarité et donc dans le cadre. De ce PLF le fait d'essayer. De mettre les enveloppes nécessaires à l'ensemble de ces demandes mais ça illustre aussi le fait que dans une nouvelle démocratie. Dans ce XXIe siècle, il serait grand temps aujourd'hui de réfléchir vraiment en profondeur sur le revenu de base, le revenu universel qui devrait assurer un socle financier un socle de solidarité tout au long de la vie que l'on soit jeune, moins jeune, ou qu'on soit âgée ou retraitée ce socle de club de base permettrait véritablement de simplifier nos dispositifs de simplifier le système qui est particulièrement complexe et il rentrerait bien dans un régime aujourd'hui de revenus globaux pour l'ensemble des populations dans laquelle dans lequel, bien sûr. La retraite devrait pleinement s'intégrer. Donc vous voyez bien que. Il s'agit bien de mettre en prospectives véritablement des réformes de fond. Et cette réforme là, je vous le redis, elle reste toujours Calais à la fin du XXe siècle. Ce n'est absolument pas une réforme d'anticipation ce n'est absolument pas une réforme de prise en compte des évolutions sociologiques. Ce n'est absolument pas une réforme de prise en compte des besoins nouveaux. Et voilà et cet article 20 même modestement dans cette prise de parole, l'illustre totalement. Je vous remercie madame Vaneck. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Avec cet article 20. Dont nous demandons la suppression se termine l'examen de votre projet de loi réformant la retraite projet inutile et injuste pour les travailleurs de notre pays les conditions par votre faute, dans lesquels nous avons traité ce texte qui va impacter de manière néfaste nos concitoyens est inédite dans notre assemblée réputé sage et attaché au travail de fond et au débat d'idées. De votre faute. Monsieur le Ministre Mesdames et messieurs nos collègues de la droite sénatoriale de votre faute et en particulier par l'activation de la procédure de vote bloqué. Nous avons dû renoncer à débattre sur nos propositions. Nombreuses et alternative, notre travail parlementaire a été foulé aux pieds les élus de la République que nous sommes méprisés. Les Français ont compris votre manoeuvre il ne le comprennent pas, ils ne la comprennent pas ils ne le pardonneront pas. Vous porterez la seule responsabilité du vote de ce texte néfaste pour eux sauf si en conscience et sur le fil. Vous vous décidez à retirer votre projet vous le pouvez encore. Merci madame la présidente. Donc nous sommes au dernier article de cette de cette réforme. Pendant 10 jours nous avons bataillé jour et nuit contre cette réforme des retraites injuste et brutale article après article nous avons démonté les mensonges du gouvernement sur la nécessité de cette réforme sur le déficit du du système de retraites sur la revalorisation des petites pensions sur le coût des régimes spéciaux face aux centaines de propositions que nous avons fait pour des financements alternatifs pour une meilleure prise en compte des carrières hachées. Pour une revalorisation des pensions des femmes pour une meilleure prise en compte de la pénible des pénibilité au travail pour améliorer le temps d'emploi des seniors. Nous avons trouvé un mur. La droite sénatoriale s'est enfermé dans le silence en refusant de participer au débat et les gouvernements dans la surdité en refusant d'écouter nos arguments main dans la main, ils se sont obstinés à bâillonner l'opposition. Usant de tous les stratagèmes possibles pour couper court au débat. Les articles 38 et 42 du règlement du Sénat qui limite le nombre d'aérateurs pour voir s'exprimer la réécriture d'articles faisant tomber plus de 1000 amendements puis l'article 44,2 de la Constitution qui autorise le gouvernement à s'opposer à l'examen de dizaines d'amendements et enfin l'arme de destruction massive du débat le 44 tiré trois au vote bloqué qui met fin à tout débat contradictoire et oblige à un vote unique sur le texte et les allant non choisi par le gouvernement face à la résistance de l'opposition, le gouvernement a dû procéder à un coup de force pour faire passer une réforme dont personne ne veut, mise à part la droite sénatoriale brutalisant le Sénat pour obtenir un vote de force. Le gouvernement a brutaliser le pays dans la rue et au Parlement. Nous continuerons de nous battre pour préserver les acquis sociaux des Françaises et des Français et pour faire échec à cette réforme illégitime. Merci madame Le Houerou. Cet article 20 ajoutent 400 millions d'euros au plafond des dépenses de l'assurance vieillesse pour l'année 2023 si ces 400 millions supplémentaires sont liés notamment à la revalorisation du minimum contributif et à la revalorisation accordée pour rattraper l'inflation cet article entérine l'ensemble de la réforme du gouvernement cet article tient compte des premiers gains attendus du report de l'âge de la retraite à l'art. Du de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Vous oubliez les multiples budgétaire négatifs de cette réforme. Selon l'OFCE. Si on cumule les dépenses induites, chômage, maladie, et les effets micro et macro économique contraction des salaires, baisse de l'activité, l'économie réalisée ton ma de 8 milliards d'euros à horizon 10 ans. Le Haut conseil des finances publiques établie qu'elle devrait coûter 600 millions d'euros. Il n'est pas en mesure d'évaluer l'incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques. Or l'incidence, la majorité des Français et des Françaises la ressentiront dans leur corps meurtri à 64 ans par conséquence la trajectoire établit dans cet article 20 et infondées en cohérence avec ce que nous avons défendu tout au long de l'examen de ce projet de réforme des retraites, c'est-à-dire notre opposition totale et argumentée à cette réforme injuste et injustifiée. Nous demandons la suppression de cet article 20, nous dénonçons ainsi le mépris envers l'opposition sénatoriale nous dénonçant le mépris du président de la République envers les syndicats qu'il refuse de recevoir, nous dénonçons le mépris envers les salariés, nous dénonçons le mépris envers les Français. Une seule issue raisonnable le retrait. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons ici le dernier article de ce texte. Si 400 millions d'euros supplémentaires sont liés notamment à la. Revalorisation du minimum contributif. On ne peut oublier en ce moment les à les approximations, voire les contre-vérités proférées par le gouvernement depuis 2 semaines sur ce minimum retraite à 1200 euros avant d'être confondu. Au terme de l'examen de ce texte. Quel bilan tristesse et colère car le choix d'un PLFSSR nous a empêché de prendre en compte, de nombreuses situations en raison des règles d'irrecevabilité d'un texte budgétaire, ça c'était l'acte Puis nous avons eu l'acte II, les articles 38 42 du règlement intérieur du sénat petit livre Vert devenus célèbres. Enfin, l'acte 3 c'est l'artillerie lourde. L'article 44 de la Constitution, le vote bloqué qui permet au gouvernement de choisir les amendements débattus. Le gouvernement voulait une victoire. Il ne l'a pas eu à l'Assemblée nationale. D'autant qu'une partie de sa majorité relative ne veut pas de ce texte. Il a eu au Sénat il a piloté le texte main dans la main avec la droite sénatoriale quand tous les moyens constitutionnels tous les moyens de nos règlements sont mis en oeuvre pour faire passer un texte dont les Français ne veulent pas quand les syndicats ne sont pas reçu par le président de la République après un mouvement social Il y a un problème démocratique que vous devrez assumer devant les Français. Osez. Oserez-vous après ça. Une CMP conclusive droit dans les bottes. Rien ne nous permet d'en douter. Quant à nous, nous nous battrons jusqu'au bout contre cette réforme.

Merci madame la présidente juste puisqu'on est au dernier article et que nos collègues LR sont pressés de faire voter cette loi. C'est pas de la provocation, c'est c'est c'est factuel. C'est des. Bon en tout cas on va voir si vous avez bien révisé. Alors combien il y a eu de manifestations historiques.

du président de la République envers les syndicats qui refuse de recevoir mépris envers les salariés et les salariés et les Françaises et les Français. Votre projet n'est pas légitime et donc il reste effectivement quelques normalement au moins un jour à quelques heures, vous savez, on a bien compris que le le compteur était sous surveillance. Dans sur le l'hémicycle à à droite en tout cas sachez une chose, c'est que Monsieur miss, vous avez encore quelques heures pour retirer cette réforme.

Merci madame la présidente. Donc cet article final augmente de 400 millions, le plafond du minimum vieillesse qui je le rappelle, s'élève à 273,7 milliards. Il entérine surtout une réforme injuste et brutale sur laquelle nous allons bientôt devoir nous prononcer dans des conditions délétère. N'oubliez pas mes chers collègues, que les Françaises et les Français nous regardent à l'heure où nous parlons des dizaines et des dizaines de courriels s'accumulent sur nos boîtes Mail Sénat a envoyé par des enseignantes et des enseignants de nos départements respectifs qui nous demandent de les entendre la plupart ce sont des femmes il et elle s'appelle Christelle Anne Julie Katiana Abdennour Sébastien Carol Florence Cindy Luc Bruno Natalie et Delphine comme tant d'autres il et elle ont consacré leur vie à l'éducation de nos enfants à faire vivre à l'école publique et laïque de la République avec courage et conviction. Malgré un contexte chaque année plus difficile lorsque leur mission ça sera achevée. Nous leur devant le droit au repos dans de bonnes conditions, voilà ce dont il est question aujourd'hui être juste simplement juste avec celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie en faisant de leur mieux c'est seul à reconnaître la valeur du travail et pas celle du capital. C'est cela la justice sociale, pilier de la République, seule garante de l'adhésion des Françaises et Français à ses principes. Car si la République est injuste et brutale avec celles et ceux qui travaillent dur, alors elle n'est plus fidèle à elle même. Voilà le choix qui est le nôtre ce soir préserver ce que nous avons de plus sacré ou prendre le risque de fissurer. Une fois de trop, le pacte républicain. Soyons à la hauteur de cet instant retirer cette réforme. Madame Meunier. Monsieur Kanner. Et à. Madame la présidente, monsieur le ministre. nous en sommes, c'est-à-dire à à la fin de nos travaux bientôt. Je voudrais vous livrer ces quelques mots qui ont été prononcés ici même. Il y a bientôt 13 années. Il s'adresser. Aux rangs de la droite diverses ici présente. Vous pouvez bomber le torse mais il y aura un autre appel, cette fois devant le peuple et c'est lui qui tranchera. Vous marquez de mauvais points. Tous les sondages le montrent les 2 tiers des Français sont opposés à votre réforme, vous devez en tenir compte. Le gouvernement se réfugie dans une position de faiblesse qui sera jugé par le peuple. Au delà des péripéties de vote de notre assemblée. On sait la réputation du Sénat sous la IIIe République. La 4ème République et le début de la Ve. Le Sénat ne doit pas redevenir la chambre noire de la République, la retraite c'est une mesure de civilisation. ce ne sont pas les salariés seuls qui doivent payer, il faut mettre le capital à contribution. Si vous ne prenait pas les mesures que le peuple attend les conséquences seront redoutables. Il faut suivre un autre chemin, le nôtre. Pierre Mauroy, face à la réforme de 2010. Mes chers collègues. Ces mots sont prémonitoire retenez-les retenez-les et pour ce qui nous concerne nous continuerons toujours en permanence à vous demander, monsieur le Ministre, de retirer votre réforme.

aujourd'hui. C'est le dernier. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le présente le présent amendement et le dernier de ce texte visait à supprimer cet article 20. Qui actait la rectification des dépenses de la branche vieillesse pour l'année 2023. Les objectifs de dépense de la branche vieillesse ont fixé à 273 7 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de Sécurité sociale contre 273 3 milliards d'euros dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Ces 400 millions d'euros supplémentaires sont principalement liées à la revalorisation du minimum contributif et à l'augmentation accordée pour rattraper l'inflation lors des débats. Nous avons présenté de nombreuses propositions pour permettre de réellement revaloriser les pensions de retraite pour l'ensemble des Français pour que nos retraités puissent vivre dignement. Vous avez fait le choix de ne jamais entendre nos propositions pourtant chiffrée. Et concrète. C'est pour cela que nous proposons la suppression de cet article que nous jugeons inadapté et voilà, mes chers collègues dans quelques amendements. Nous y sommes. Ah, là nous sommes à la fin de cette réforme de régression sociale. Je tenais à saluer l'attitude de l'ensemble des groupes de gauche qui ont su dignement représenté les 70% des Français opposés à cette réforme et les millions de personnes qui se mobilisent dans la rue pour dénoncer les conséquences de cette réforme. Ensemble, nous aurons pu assister aux premières loges à la confirmation de l'alliance entre la droite et la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron qu'ils seront particulièrement qui se seront particulièrement bien entendu pour utiliser l'ensemble des points du règlement pour contrevenir au droit parlementaire. La fin de l'examen de ce texte n'aura malheureusement pas été à la hauteur des attentes des Français. Mais nous continuerons inlassablement à défendre la justice sociale pour nos concitoyens. Merci madame la présidente. Et quoi après. Des millions de personnes manifestent. On n'a jamais raison sans le peuple. Et encore moins contre lui. Donc, ce texte va être adopté par notre chambre, il a été rejeté à l'Assemblée nationale. Nous avons débattu ou plutôt soliloque pendant toute la première partie. Vous avez voté nuitamment l'article 7. Et puis la belle machine feutrée du Sénat s'est déréglé. Tous les articles de réduction de la capacité d'intervenir. Des oppositions ont été mises en oeuvre. Nous allons voter ce soir et demain. Demain une CMP 7 sénateurs 7 députés vont adopter un texte qui sera rejeté par 70 à 80% des Français selon les âges qu'on considère et après, chers collègues. Et après si la démocratie se fait sans le peuple. Qu'est-ce qu'il y aura après. Et nous serons tous ceux concernés par ce qui viendra après. qui viendra après. Madame Cohen. Oui merci madame la présidente. Cet article 20 prévoit les dépenses j'apprends branche assurance vieillesse censé justifier la réforme des retraites, discutée depuis 10 jours, ici au Sénat. Cet article permet de constater que l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans et l'âge légal de départ en retraite à 64 ans aura pour conséquence d'ici 2026, de réduire le déficit. Soit disant de 15 7 milliards à 14,9 milliards d'euros. Ainsi donc non seulement votre réforme est injuste pour les Françaises et les Français qui vont devoir travailler deux années supplémentaires impopulaire puisque 80% d'entre elles et opposés sont opposés à cette réforme mais également inefficace puisque le déficit du système des retraites demeure. C'est pourquoi nous demandions un amendement de suppression pour notre part, nous proposons une réforme pour un droit à la retraite à 60 ans avec une pension à taux plein garanti pour une carrière complète avec prise en charge de cotisations pour les périodes de travail, y compris les périodes de chômage, de formation des études du congé parental maladie invalidité. Un projet alternatif plus juste qui tient compte de la pénibilité des carrières longues. C'est possible, ce serait possible si on faisait le choix d'augmenter la cotisation des employeurs en mettant à contribution les revenus financiers des entreprises en donnant aux salariés de nouveaux pouvoirs d'intervention dans les entreprises en augmentant les salaires garantissant l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Conformément à la loi, le gouvernement et la majorité sénatoriale nous disent, enfin des 35 heures 43 années annuités 64 ans nous répondrons que pour nous c'est 32 heures 37 donc retraite de retrait de cette réforme illégitime qui est injuste et inutile, écoutez la voix des Françaises et des Français. Écoutez les voix majoritaire qui s'élève dans le pays. Stop au mépris. Le président de la République doit recevoir les syndicats et vous devez abandonner ce projet n'efface.

et on voit que le solde par rapport au PLFSS 2023 a été dégradé de 300 millions d'euros. Et je dirais presque, tant mieux, tant mieux, c'est la traduction des dépenses supplémentaires liées à faire en sorte que des mesures sociales soient prises à travers de l'effort supplémentaire qui est demandé aux Français et notamment effectivement c'est une dégradation du solde liés notamment à la revalorisation des petites pensions à travers le minimum contributif le Mico, mais également à travers la réévaluera revalorisation de la PMR le minimum pour les. Les agriculteurs. Donc on voit bien que quand on prend. Des dispositions qui font en sorte qu'on va vers un rééquilibre de notre système de retraite avec derrière des recettes supplémentaires. Il faut faire en sorte de prendre un certain nombre de mesures sociales, elles ont une répercussion immédiate quant la répercussion de l'augmentation des recettes et plutôt plus tardive c'est la raison pour laquelle plus on tarde à prendre des décisions. Monsieur le Ministre et plus la réforme elle est difficile. C à fait 4 ans que l'on propose ce type de réforme justement sans prendre de retard pour faire en sorte que on arrive à l'accompagner de façon beaucoup plus facile. Néanmoins, pour 2000 des 23, le solde sera encore de moins 3,9 milliards. En ce qui concerne la branche vieillesse et on voit bien que ce solde, continue à se dégrader au fil des temps, surtout si on ne prend aucune mesure compensatoire et il se dégrade. Je vous le rappelle, mes chers collègues, avec une démission une diminution de pouvoir d'achat de nos. Retraités puisque le niveau moyen des retraites va en diminuant dans les trajectoires que l'on a déjà étudié notamment à travers le En ce qui concerne cet équilibre. Nous avons l'homme a effectivement proposé un, un, un choix difficile. Aux Français. Un choix qui effectivement demande un effort collectif, c'est la raison pour laquelle les mesures sociales d'accompagnement. pour le plus grand nombre parce que la réforme Touraine c'est pour ceux qui commencent tôt le décalage de bornes c'est pour ceux qui commencent tard donc la réforme du mélange des deux est une réforme plus équitable la réforme déjà j'anticiper ces pots. Permettez madame c'est pour prendre en compte effectivement les usure professionnelle les accompagnements que nous avons proposé dans la commission, notamment à travers la recette. La retraite progressive ou à travers l'incapacité permanente, prix des 60 ans sont des mesures qui adoucissent effectivement l'usure supplémentaire qui peut être traduites dans des métiers difficiles compte tenu de l'effort supplémentaire que nous réclamons mais que faire quand vous avez un système par répartition, il y a pas 36 solutions là déjà on l'a déjà largement défini quand vous avez un nombre de cotisants qui baisse une durée de retraite qui dure de plus en plus long. les Français comprennent bien qu'il faut quand même faire quelque chose et c'est simple, si on ne propose pas. Si on ne propose pas effectivement cet effort collectif aux générations d'aujourd'hui, ce seront les générations suivantes qui le paieront et si vous ne faites pas ça, le système est simple et vous le savez bien, vous le savez bien. Ça veut dire quoi une augmentation des cotisations, c'est une baisse du pouvoir d'achat pour ceux qui travaillent. Une baisse des retraites, c'est une baisse, une baisse des pensions, une baisse des pensions situe. Une baisse du pension c'est une baisse du pouvoir d'achat pour les retraités. Est ce que vous pouvez laisser séquence. Ne remportèrent poursuivre s'il vous plaît. Depuis plus de 4 ans. Nous l'avons dit, nous ne souhaitons pas faire des retraités pauvres. C'est la raison pour laquelle nous assumons nos responsabilités pour faire en sorte que l'on propose un système qui certes. Est un effort on le reconnaît bien volontiers mais qui est tout à fait nécessaire pour faire en sorte que l'on puisse équilibrer ce système et donner confiance à nos jeunes. Mais l'affaire n'est pas fini. L'affaire n'est pas fini, Monsieur le Ministre. Puisque j'espère un vote bien sûr positif. De notre assemblée et nous allons attaquer la phase suivante de la CMP sachez Monsieur le Ministre. Que nous avons travaillé largement ce texte propos. Pour proposer des mesures d'adoucissement et ça. Mais Madame. Ah ça si c'est à moi, en tant que rapporteur membre non madame rapporteur. Je suis membre de la majorité sénatoriale. Ça n'a échappé à personne mais en tant que rapporteur, je serai membre de la CMP. En tant que rapporteur membre de la CMP. Je me permets, n'en déplaise à certains. De m'adresser à monsieur le ministre pour lui dire que nous serons fermes sur les propositions que nous avons proposé par rapport. Ce sont des propositions de justice sociale qui sont indispensables pour la pour l'adoption de ce texte. Je tenais à vous le dire devant vous toutes et vous tous car c'est une affaire d'importance. Merci. Merci madame la présidente, là l'avis est défavorable, toujours comme depuis l'article 14. Parce qu'il s'agit de d'articles qui sont obligatoires, si on veut que le PLFSS soit recevable, il y a un certain nombre de règles organique qui détermine les articles obligatoire et le contenu obligatoire d'un PLFSS, qu'ils soient actifs qui peut rectificatif au initial et donc la vie par définition défavorable. Je voudrais simplement ajouter 2 remarques, la première c'est que la dégradation du solde qui apparaît dans cet article est le signe tangible illustration tangible des effets des premiers effets en 2023 de la mise en oeuvre de la réforme que nous vous proposons d'adopter, c'est. Parmi les premiers signes tangibles et plus important de l'impact des conséquences que le texte que nous vous proposons d'adopter peut avoir. Ah et et j'espère aura bien sûr sur les comptes sociaux de l'année 2023 et c'est donc en un des éléments qui. Nous permet. Et qui nous a autorisés à faire le choix d'inscrire les mesures que nous portons dans le cas d'un projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif puisque nous trouvons la la trace très directe, comme dans les autres tableaux d'ailleurs. Des mesures que nous vous proposons d'adopter la la 2ème remarque que je voulais faire tiens au débat qui s'est ouvert à l'occasion de la présentation des amendements de suppression et si j'ai bien entendu de la. France de monsieur rapporteur sur la question de l'équilibre financier. le gouvernement et c'est la dernière intervention que je ferai très certainement sur les tableaux financiers et Jean saisit donc l'occasion. Le, le gouvernement souhaite à la fois mener une réforme qui permet d'améliorer le système de retraites, nous pouvons avoir. Des divergences mais ce que j'ai noté des différents débats. C'est qu'en matière de pensions minimum de pénibilité d'aménagement des carrières longues d'emploi des seniors d'attribution de droits que beaucoup ont qualifié de mesure juste je pense sapeurs-pompiers. Je pense aux orphelins. Je pense aux possibilité de rachat de trimestres. la difficulté qui peut apparaître ou de la divergence qui peut apparaître entre nous n'est pas une divergence d'opportunité mais une divergence de curseur sur. La possibilité d'en faire trop de n'en faire pas assez sur ces points là il y a un autre aspect sur lequel il y a une divergence très clair, c'est comment est-ce que nous assurons l'équilibre du système. Nous avons fait un double choix. Du premier choix c'est l'équilibre. C'est le retour à l'équilibre en 2030 parce que nous considérons que le meilleur service à rendre aux générations qui viennent et finalement le principal acte de solidarité, c'est de garantir l'équilibre du système et. J'ai en tête les mots que j'ai prononcée dans la discussion générale sur le texte. Toutes les responsabilités que j'ai eu l'honneur d'exercer toutes les expériences que j'ai vécu et chacune des fonctions que j'ai eu à, à remplir mon convaincu que l'équilibre financier. La discipline budgétaire sont les conditions de l'action et ce sont les conditions de l'action et des priorités politiques que nous pouvons avoir et donc ce 1er choix c'est l'équilibre et le 2ème. C'est atteinte cet équilibre sans remettre en cause la politique de compétitivité que nous menons depuis maintenant de nombreuses années, qui je crois en terme d'emploi d'attractivité et de redressement industriel porte ses fruits et sans toucher au pouvoir d'achat des Français, qu'ils soient cotisants aux bénéficiaires des retraites. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix du travail et c'est comme cela que nous avons construit l'équilibre budgétaire de ce système et c'est aussi une des raisons qui m'amènent à confirmer l'avis défavorable du gouvernement sur cette série d'amendements. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant passer aux dernières amendement de du projet de loi et le dernier amendement est un amendement de Madame Poncet Monge. Qui sera défendue par Monsieur

qui va même au-delà du texte au-delà du dernier article soit écrit par ma collègue Raymonde Poncet Monge qui avaient envie qui avait vraiment envie débat de ce texte qui avaient déposé des amendements sur tous les articles et que vous avez frustrés vous avez frustrés son envie de débattre, notre envie de débattre. D'abord en choisissant ce véhicule législatif avec un temps contraint on va le redire ce temps contraint qui était déjà un 1er signe de votre fébrilité par rapport à votre. À votre réforme qui au cours au cours des discussions vous avez peu à peu éteint le débat. D'abord, puisque la droite sénatoriale a fui le débat sur l'article 7 a fui le débat sur le report de 62 à 64 ans. La mesure la plus brutale, le coeur de cette réforme vous avez déserté le débat, vous avez par une manoeuvre parlementaire fait tomber les amendements de la gauche et vous nous avez contraint à ne pas en parler et puis vous avez au fur et à mesure encore plus contraint le débat quand on avait commencé à démontrer l'inefficacité la faiblesse des mesures d'atténuation de la brutalité de la réforme cette fois-ci c'est le ministre qui a dégainé le 49 3 sénatoriale pour ne pas que nous puissions en débattre. Alors vous allez sûrement

avec l'ensemble des syndicats au mépris au mépris des millions de travailleurs puisque on va le redire 9 travailleurs sur 10 sont hostiles à cette réforme et vous les avez ignoré. Vous avez brûlé tout au navire. Monsieur le Ministre votre seule bouée de sauvetage était ici la droite sénatoriale. Une des droites les plus conservatrices du pays qui vous a accordé. Son vote ici au Sénat, mais votre réforme était non nécessaire injuste et brutale. Nous continuerons de le dire, les travailleurs continueront de le dire le pays continuera de le vous le dire, jusqu'au retrait. Je vous remercie. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président, puisque ça n'a pas été fait, je vais me permettent de présenter l'amendement. Il y Il y a une aversion des rôles. Donc l'amendement précisé que la présente loi ne s'applique pas dans lesquels dans les collectivités d'outre- mer. La commission n'a pas retenu. Effectivement ce ce type de raisonnement car nous pensons. Que loi de la République doit s'appliquer dans tous les territoires. On doit certes. Considérer les différences qu'il peut y avoir, notamment avec nos amis des Outre-mer et nous ne les avons pas oubliées à travers ce dispositif puisqu'on a pris un certain nombre de mesures concernant Mayotte concernant des revalorisations et concernant également. La différence. Qui existait déjà dans le recours sur succession en ce qui concerne l'ASPA grâce à Viviane Malet cela fera partie encore de de discussion. Monsieur le Ministre, je tenais à le souligner, nous n'oublions pas nos à 3 maire néanmoins avis défavorable par rapport à à votre proposition. favorable. Avis du gouvernement. Avis défavorable. Attends, mes chers collègues. Nous allons procéder au vote unique. Sur le texte. En application de l'article 44 dernier alinéa de la Constitution. Et de l'Arctique 42 alinéa 9 du règlement du Sénat. Le gouvernement a demandé au Sénat de se prononcer par un seul vote. Sur les articles 9 à 20. En ne retenant à partir du moment où cette demande a été formulée. Que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Sans remise Sans remise en cause des amendements précédemment adopté à l'article. Mais aussi sur l'ensemble du texte. Monsieur le Ministre. Contre tenu des retraits d'amendements intervenu. Et pour la clarté et la sincérité de nos débats et de notre vote. Pouvez-vous nous rappeler la liste des amendements et sous-amendements acceptés par le gouvernement. Je vous donne la parole. Merci monsieur le président. Voici donc la liste des amendements et des sous-allemand des sous-amendements acceptés par le gouvernement dans le cadre du vote unique en application de l'article 44 dernier alinéa de la Constitution. Et de l'article 42 alinéa 9 du règlement du Sénat.

Pour les amendements portant additionnel après l'article 10, les amendements numéro 22 95 20 24 21 61 rectifié bis. 45 47 400 ce Pour l'article 11, les amendements 24 88 rectifier bis et 21 62. Pour les additionnel après l'article 11 l'amendement 1904 rectifié bis à l'article 12 l'amendement 21 63 21 64 et 21 65.

Pour les additionnel avant l'article 14 l'amendement 25 63 rectifier. À l'article 14 amendements 47 23 à l'article 15 47 24 et l'article 16 21 84 ainsi que tous les amendements identiques et à l'exclusion de tous les autres, y compris des amendements portant articles additionnels. Je précise Monsieur le Président, qu'en comparaison avec la demande formulée vendredi matin. Le gouvernement ne retient pas les amendements 21 41 et 20, 21 45 sur l'article 9, car ils auraient été entre-temps retirée par leur Par contre ils sont inclus les amendements 46 50 sur l'article 10 et 47 57 sur l'article 13 qui sont des amendements de coordination présenté par le gouvernement et que je n'avais pu présenter lors de la première déclaration de vendredi matin. Merci, monsieur le Ministre, en application de l'article 42 alinéa 5 de notre règlement et conformément à la décision de la conférence des présidents lors de sa réunion du mercredi 8 mars. Je vous rappelle que les explications de vote sur l'ensemble de ce projet sont limitées à un orateur par groupe politique pour une durée de 7 minutes chacun. Et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Pour une durée de 3 minutes je vais maintenant donner la parole pour explication de vote tout d'abord pour le groupe les républicains au président Bruno Retailleau. À Cessieux.

Monsieur le président. Messieurs les Ministres, chers collègues. Enfin, nous y voilà. C'est la fin de ce marathon. Nous voilà parvenu au terme de cette course législative. À cet instant que nous croyons, il y a quelques jours encore inaccessible. Nous voilà parvenu à cet acte. Le vote qui fonde. La légitimité du Parlement, notre raison d'être. Et je le pense aussi notre honneur. Et pourtant, chers collègues de gauche vous avez tout fait pour empêcher cet acte fondamental par l'obstruction. Par l'obstruction. Plus de 8000 amendements. Et de sous-amendements. Des rappels au règlement en veux-tu en voilà. Vous avez été recherché dans notre règlement toutes les techniques qui permettaient d'empêcher d'empêcher le vote. Vous étiez mauvais perdant puisque vous aviez par avance anticipé votre défaite. Et c'est la raison pour laquelle vous vouliez empêcher le vote, mais nous y voilà, et ce vote sera pour nous déjà. Une victoire, mes chers collègues, mes chers collègues. Cette. Obstruction. Nous a permis d'entendre énormément de prise de parole de nos collègues de gauche sans qu'on sache bien qu'elle s'était vos propositions, vos solutions.

Que la France va devoir dans les prochaines années. Affronter l'autre choc il y a bien sûr le choc climatique mais il y a aussi le choc démographique du vieillissement. Les départs en retraite, vont être multipliés par 4 par 5. Que faisons-nous. Que voulez-vous faire. Nous, nous agissons. Nous avons voulu agir et cette réforme, nous l'avons voulu, Monsieur le ministre, messieurs les Ministres, mais Monsieur le Ministre Dussopt tout particulièrement. Je voudrais m'adresser à vous. Vous irez porter ce message au président de la République, cette réforme nous allons la voter. Mais nous ne votons pas pour lui. Cette réforme. Nous la votants parce que c'est notre réforme c'est ici qu'elle est née. Nous la voterons parce que nous l'avons modifié c'est notre texte que nous allons voter la surcote pour les mères de famille. Les orphelins, handicapés. La lutte contre la fraude. L'emploi. Des seniors qui sont souvent trop souvent à l'âge de 57 ou de 58 ans au chômage. Les questions de la pénibilité de mesures professionnelle. Ce sont ces ajouts que nous avons voulu apporter à ce texte là. Si nous votons cette réforme ce n'est pas parce que le gouvernement des mails Macron la propose. Non c'est pour l'intérêt national. Parce que nous voulons. Sauvegarder un régime de retraite par répartition. J'ai entendu les moqueries. Sur les questions de chiffres et d'équilibre. Non ce qui se moque des chiffres se moque des Français derrière les chiffres, il y a des déficits derrière les déficits. Il y a l'argent des Français et derrière l'argent des Français. Il y a la peine des Français. Le régime. Par répartition que nous soutenons. C'est celui qu'il faut sauver parce que demain sinon il y aura un effondrement du pouvoir d'achat de nos aînés et nos jeunes devront payer 2 fois la retraite notre votre retraite et leur propre retraite. C'est cela que nous voulons évidemment préservée, comme nous voulons préserver la croissance de demain qui est le chemin de la prospérité et derrière cette réforme, il y a le taux d'emploi il y a cette capacité que nous aurons de mettre encore plus de travail dans l'économie française. Nous sommes le dernier un des derniers pays européens par la quantité de travail et c'est l'appauvrissement assuré si nous en restons là nous voulons ce chemin de croissance chemin de prospérité. Vous voulez la décroissance, le déclassement et l'appauvrissement, mais au-delà de ces considérations. Matériel. Nous nous battons pour quelque chose de beaucoup plus sans ciel que les retraites ou la croissance. Nous nous battons aussi pour des conditions immatériel. Nous nous battons, parce que derrière cette réforme, derrière ce régime Inter générationnel. Il y a un lien. Il y a ce lien entre les générations, qu'exprime le régime par répartition et c'est ce lien qui nous manque tant en France, dans une France archipel lisez morcelé fracturé qui matérialise que nous sommes un peuple, une seule communauté nationale, voilà pourquoi nous allons. Monsieur le Ministre, Mesdames, messieurs, mes chers collègues la voter et je terminerai par des remerciements remerciements d'abord. Au rapporteur au rapporteur à la rapporteure générale qui a fait preuve d'une grande combativité. rapporteur à notre rapporteur René-Paul Savary avec son énorme travail. Avec sa zénitude même si sous les attaques de la gauche. Bravo. Chers collègues. Notre président de commission dont la voix. Haut perché se transforme parfois en lames coupantes. Et certains ne savent ici et en en fait les frais. Merci Je voudrais aussi remercier nos collègues qui ont été présents, regardez cette présence encore merci mes chers collègues d'avoir enduré des séances. Qui n'apportait souvent rien aucune solution. Mais où il fallait faire face aux manoeuvres d'obstruction des oppositions merci mes chers collègues, monsieur le président, enfin je voudrais terminer. Une fois n'est pas coutume, parce que je ne pense pas que dans l'histoire récente du Sénat. Notre administration nos services aient été autant mis à l'épreuve. Je ne parle pas de la quantité d'arbres qui ont dû être abattus pour être transformé en sous-amendement. Je parle du travail. Je parle du travail de l'administration du Sénat qui est aussi notre honneur qui a montré dans des moments extrêmement tendue. Difficile qui a toujours tenu qui a joué son rôle de conseil parce que pour nous, c'est fondamental. Je veux parler bien sûr du secrétaire général de la séance mais aussi de. Tous les collaborateurs et je vous propose. Précisément, mes collègues pour terminer ce marathon de vous lever et de les applaudir.

La parole est à notre collègue Monique Lubin s'exprimer pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.

Monsieur le président. Messieurs les ministres, madame la présidente de la commission des affaires sociales. Madame et monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Je vais moi aussi. Commencé par remercier. Tous ceux qui ont travaillé sur ce texte effectivement très important. De cette mandature. Nos collègues. Rapporteurs bien évidemment. Madame la présidente de la commission. L'administration dans son entier. Tout ce que l'on voit tout ce que qu'on le que l'on ne voit pas et bien évidemment nos nos collaborateurs soyez remerciés de ce travail extraordinaire de ce travail de fond pour ce qui fut en effet un marathon. Cette journée, messieurs les Ministres, Mesdames messieurs restera une journée noire. Pour tous les salariés de ce pays. Nous savons que vous voterez le recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Parce que nous savons, chers collègues, que vous avez négocié avec le gouvernement. Pour voir aboutir ce que vous attendez depuis si longtemps. Parce que nous savons, messieurs les ministres, que le gouvernement s'est soumis. Afin de s'assurer le vote majoritaire du Sénat. Dont vous avez impérativement besoin pour apporter un minimum de légitimité à votre texte. J'irai droit au but. Vous avez voulu faire peur aux Français en leur disant que les régimes de retraite était en faillite et c'est faux. Si c'est faux. Votre réforme est une réforme idéologique. Vous n'avez jamais été favorable aux mesures qui permettent aux salariés de ce pays de vivre mieux. Vous n'avez pas aimé la retraite à 60 ans. Vous n'aimez pas les 35 heures.

Elle était injuste parce qu'elle concerne essentiellement les salariés les plus proches de leur départ à la retraite, ceux qui travaillent depuis longtemps ce qu'il a exercé les métiers les plus difficiles, ceux qui perçoivent la plupart du temps les salaires les plus modestes. Elle est brutale parce qu'elle prend effet immédiatement, dès septembre 2023. Aucune réforme depuis celle de 1982 ne s'est appliqué immédiatement. Autrement dit, à des salariés dont le départ à la retraite et prêt. Ou en cours de préparation, aucune réforme des retraites n'a jamais été aussi brutale dans ce pays. Elle est brutal pour les salariés qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans. Parce qu'il y aura bien un report à l'âge de 62 ans. Malgré tous les éléments de langage que vous avez déployés pour infirmer cette donne. Elle est inéquitable parce que les seuls efforts vont porter sur les salariés. Rien n'est demandé aux employeurs au prétexte que nous serions déjà trop exigeant avec les entreprises de ce pays en termes de cotisations sociales et d'impôt. Pourtant depuis 5 ans les cadeaux fiscaux et sociaux pleuvent sur les entreprises à un niveau jamais connu en France. Elle est brutale. Elle est brutale. Dans sa totalité et pour vendre votre projet de loi. Vous avez essayé. De nous conter des histoires. Et je mesure mes mots. Vous savez ils essayaient de nous de nous vendre. Que les femmes y trouveraient leur compte que les femmes seraient les grandes gagnantes de cette réforme. Il n'en est rien. Et cela a été démontré immédiatement, c'est tellement faux. Que la majorité vous arrachent un bonus pour compenser la perte de bénéfices des droits familiaux qui s'imposera aux femmes, mères de famille et qui devront travailler 2 ans de plus. Vous avez aussi essayer c'est presque encore plus grave, c'est au moins aussi grave. De nous faire croire que tous les salariés qui ont eu de retraite complète aurait un minimum de retraite à 1200 euros brut. Ça n'est pas le cas, ça a été démontré. Nous avons mis eut même droit à des excès de langage. De certains ministres qui annonçait deux millions de bénéficiaires là où on se rend compte aujourd'hui que ça sera bien moins que ça. Elle est brutal avec les seniors dont tout le monde sait qu'ils rencontrent les plus grandes difficultés à retrouver un emploi. Ils verront leur situation se précariser d'autant plus que vous avez imposé il y a peu une diminution des droits au chômage. Et puis, chers collègues, je ne vais pas passer sur la manière dont vous avez que vous avez eu d'aborder ce texte. Vous avez été quasiment mutique durant toute la durée de son examen. Nous avons fait des dizaines et des dizaines de propositions, aucune n'a mérité que vous vous y intéressiez. Vous avez refusé le débat et, en le refusant vous avez manqué de respect à tous ceux qui vont subir les conséquences de ce report et qu'qui voulait entendre vos arguments. Vous avez certes apporté quelques nuances pour faire croire que vous vouliez adoucir un peu la brutalité de ce texte. Mais la vérité c'est que vous vouliez le durcir encore plus en proposant un amendement. Monsieur le Président, Retailleau qui revenait sur la clause du grand-père. Instaurée par ce projet de loi c'est-à-dire supprimer les régimes spéciaux avec effet immédiat. Vous n'êtes pas allé au bout, parce que vous risquez d'être mis en minorité. Et ça aurait sacrément de permis. Votre éventuelle victoire. Et que dire enfin de l'attitude du président de la République. Qui refuse obstinément de recevoir les organisations syndicales. Après des semaines de protestation. Le peuple gronde. Et le président de la République regarde ailleurs. Cela me fait penser à ce qu'avait dit un autre président de la République. Celui. Celui qui nous avait donné la retraite à 60 ans. Celui qui avait amené des changements extraordinaires dans les années 80 pour tous les salariés de ce pays, celui qui nous avait prévenus que vous toucherez aux retraites que vous touche riez à la protection sociale que vous vendriez tout au privé. Nous aurions dû l'écouter. Mais cette phrase reste désormais marqué en août, le président de la République actuel n'écoute pas le peuple, le peuple s'en souviendra. Pour le Je vais donner la parole Pour le groupe de l'Union centriste. Notre collègue Olivier Henno. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, madame la présidente de commission madame mesdames messieurs le les rapporteurs ça nié. Alors va tuer le suspense majoritairement très majoritairement notre groupe votera ce ce texte. On lui est. Un peu fatigué d'avoir. Travaillé un peu fatigué aussi de. Vous avoir écouté mes chers collègues. Mais on aborde cette. Fin de discussion sans regrets sans remords avec une sérénité, un soulagement. Un soulagement pour la place et la crédibilité du Sénat. Un soulagement pour notre système de retraite par répartition. Un soulagement pour. La démocratie représentative. Voilà, nous sommes au bout du texte comme nous vous l'avez dit le président. Vous n'avez pas été pris par surprise, c'était un engagement qui avait exprimé le sénat et son président et il a été Capitaine dans la tempête, le Sénat et son président et la majorité ça sénatoriale ont tenu leur objectif. Je veux remercier à mon tour. Les présidents de groupe pour l'organisation des débats, les rapporteurs un formidable. En argumentation ayant travaillé faisant notre fierté. Débatteur infatigable. Ça lui aussi les groupes d'opposition. ils ont fait le choix de la flibusterie. Disons-le, c'est une flibusterie de notable. Ça ne va pas forcément vous faire plaisir, mais c'est ainsi. Mes chers collègues. Alors ce texte. Ce texte. Il mérite pas l'indignation que vous lui avait prêté, il mérite pas non plus un enthousiasme excessif. Ça n'est pas la mère des réformes, mais il a une utilité une exigence morale. Pour les jeunes générations une utilité. Parce que c'était nécessaire. Lire un texte. Il n'y a pas d'alternative de nouveaux efforts notamment des départs à la retraite plus tardif devront être réalisés afin de pérenniser notre système de retraite. Je vais répéter. On a beaucoup écouté ce matin on sont là rien lâché rien lâché rien lâcher, on revendique à notre tour le droit à la répétition. Et la répétition, c'est l'art de la pédagogie. Alors il n'y a pas d'alternative de nouveaux efforts notamment des départs à la retraite plus tardif devront être réalisés afin de pérenniser notre système de retraite. Quel est cet auteur un affreux réactionnaire un conservateur ah rétrograde. C'est un nom qui sonne à vos oreilles. C'est Pierre Moscovici. Mes chers collègues. Hein. Pierre Moscovici et donc et lui revendique l'héritage de la social-démocratie. On a entendu beaucoup de bêtises parfois sur cet. Dans cet hémicycle mais je crois que là tout à l'heure on a touché le fond, pardonnez-moi l'amour des chiffres. Ne peut pas faire bon ménage avec l'amour des gens. Alors là, excusez-moi, j'ai entendu ça tout à l'heure. Voilà la responsabilité c'est qu'elle c'est l'amour des chiffres et c'est l'amour des gens et je pense que. Vous avez cité Pierre Mauroy, si Jacques Delors avait entendu que l'amour des chips étaient. Incompatible avec l'amour des gens, je pense qu'il aurait agi dans cette assemblée, c'est un soulagement pour notre système de retraite. Un soulagement pour les retraités, parce que évidemment il y a ceux qui manifestent. Mais il y a aussi. Minorité majorité je sais pas silencieuse. Les retraités qui, après le vote de ce texte sont sécurisés par rapport à leur retraite, et par rapport, on risque qu'il pouvait y avoir sur la baisse des retraites. Les jeunes qui vont pas devoir payer 2 fois une double peine payer leur retraite mais aussi payer la dette parce que qu'est-ce qu'il a de plus irresponsable que de payer les dettes à crédit, nous ne faisons pas ce choix. Du paiement des dettes à crédit c'est irresponsable. Ce texte, ça a été dit il y a des avancées. Les seniors le CDI seniors bien sûr que le travail plus longtemps pour les seniors. C'est la clé. Ça a été dit par Élisabeth par René-Paul la question des familles des carrières longues, la politique familiale. La question de l'égalité. Femme. Les TUC, chers collègues. Il faudra pas en n'ayant pas voter ce texte revendiquer des avantages ou une justice pour les étude les pompiers. Mes chers collègues. Et puis les élus hein. Grâce à Sylvie Vermeillet. Les maires et les élus pourront et c'est pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Plus moi pourront racheter des trimestres pour les élus qui gagnent moins de 1008. 130 euros par mois mais ce texte n'est pas un chèque en blanc. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra aborder la question de la justice bien sûr ce serait cette réforme de des retraites ne peut pas tout, la question du sens du travail on n'est pas acharné. On croit à la valeur travail mais bien évidemment il faut la qualité de, de, de vie au travail, il faut la formation tout au long de la vie, il faut travailler sur l'autonomie il faut une grande loi travail nous sommes partisans de cette grande loi travail et puis. Il faut un dialogue. Social. Et ça nous y tenons beaucoup à un paritarisme rénové refondé et c'est la raison pour laquelle avec Hervé Marseille nous demandons l'ouverture le plus vite possible d'une conférence sociale et puis soulagé. Par. Et pour la démocratie représentative. Les institutions de la Ve sont solides. Tant mieux. Mes chers collègues parce que sans ces articles on y serait pas arrivé. Vous savez Aristote disait la politique c'est la rhétorique mais c'est aussi l'action et la délibération et donc l'obstruction parlementaire. C'est une impasse. Ah encore un affreux réactionnaire, c'est Laurent Berger qui dit ça. Alors il y aura un avant et un après. On a entendu un avant et un après. Mais. Oui mais surtout dans vos sur votre banc on a cité tout à l'heure, Alfred Jarry, les voraces et les Curiaces. Eh bien oui, mes chers collègues, les voraces ont battu les coriaces comme dans Alfred Jarry. Mais c'est la gauche radicale, qui a écrasé la social-démocratie dans vos rangs. Voilà la réalité de ce débat et c'est en ça que plus rien ne sera pareil. On a eu donc une gauche rassemblée sur le. Plus fautif dénominateur commun, celui de la radicalité. je voudrais citer Charles de Gaulle, la politique la plus coûteuse, mes chers collègues, la plus ruineuse pour le peuple, c'est d'être petit, hé bien cette citation, je vous l'envoie en cadeau, le Sénat se renforcer les institutions sont solides. La démocratie représentative est plus crédible et nous sommes fiers les uns et les autres d'appartenir à cette majorité sénatoriale. Je vous remercie. La parole est au président François Patriat pour le groupe il au Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Avait la parole moi je je. je. Je le président. Messieurs le ministres messieurs les rapporteurs. Madame la présidente, chers collègues. Le choix que nous allons opérer ce soir est un choix de responsabilité et un choix d'efficacité. Inutile d'être. Vindicatif agressif ou Cali caricatural. Il y va de l'avenir des générations futures. Il y va de l'équilibre et le système sociaux demain. Je voudrais dire ici que notre assemblée. Monsieur le Président, a redonné de la noblesse au débat au débat démocratique sa noblesse à la fois de débattre. Le temps qu'il a fallu trois écoutez le temps du débat mais aussi la noblesse de décider. Parce qu'une Assemblée qui débat sans vote au bout s'auto-immunise ou s'détruit par rapport à son rôle initial. comment s'est déroulé le débat. Mes chers collègues s'est déroulée en 2 mi-temps sportif comme vous. Première mi-temps du deux au sept. Pendant cette première temps chacun puisse s'exprimer longuement. Je vous rappelle que ce débat a donné lieu à presque 5000 amendements à 10 jours de débats du sans précédent sur le débat sur les retraites, les trois débats retraites qui ont eu lieu jusqu'à présent se dérouler dans un climat plutôt serein ou l'opposition souhaitait montrer son soutien à la rue au débat syndical par ailleurs est arrivé à ce débat. Première mi-temps qui se dérouler avec une multitude d'amendements de. Non je me souviens sur l'article liminaire 52 prises de parole, les unes, les mêmes que les autres pour pouvoir. Faire supprimer cet article liminaire, je m'en souviens. Inutile de de. Et puis. À partir du 7 la 2ème mi-temps, les masques sont tombés. et parce que sont tombés parce que la volonté de l'opposition n'était pas temps de débattre ce qu'elle a affirmé voulu pendant des jours et des jours, mais la volonté de l'opposition était de faire en sorte que nous ne puissions pas voter et vous l'avez dit clairement, vous l'avez dit clairement dans cette assemblée, dans les couloirs et dans les réunions des présidents, vous l'avez dit ne pas voter. Pourquoi. Pour tenter de légitimer un texte. Votée par le Parlement. Or, à qui appartient la la légitimité dans ce pays la légitimité elle appartient au Parlement. Elle appartient pas à la rue. Il faut dire ce que vous voulez, c'est le Parlement qui décide aujourd'hui et vous savez d'affronter la rue c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de de de voter des textes impopulaire. C'est pas toujours facile d'appeler à l'effort. C'est pas toujours facile d'appeler à la raison. Il y a des gens ici qui ont pris leurs responsabilités qui l'ont fait Le choix de la responsabilité de la. Et de l'efficacité. Nous l'avons fait il y a-t-il eu un bâillonnement chers collègues chers collègues nous avons écouté et vous nous reprochez parfois d'avoir été muet,

À quel moment qu'a méprisé. Qui est-ce que par le fait que sur un texte de loi annoncé aux Français travailler depuis des mois décider demain en quoi les. Le président de la République ne méprise pas les syndicats.

Un texte qui est débattu depuis 4 ans ici et en dehors de cette assemblée avec des rencontres avec tous les syndicats. Un débat qui a été menée au fond par le ministre ici présent par madame, la Première ministre avec les syndicats pour aboutir à des avancées notoires, que les syndicats ont reconnu en privé mais n'ont jamais voulu. Accepter en public par ailleurs jamais et ça a été fait, donc il n'y a pas eu de brutalité. Il y a eu un texte et moi je rappelle ici, quitte à vous faire crier ou vous faire maintenant vilipendé je trouve que ce texte il est à la fois nécessaire et protecteur. Et d'ailleurs les Français ne s'y trompent pas quand ils disent aujourd'hui à 8, pour aller vite pour dire ce qu'il pense que le texte sera voté. Ça n'est pas par notre entêtement parce qu'ils savent très bien, on est même que ce texte il est nécessaire pour assurer la survie, la survie du service, pour demain et ils le savent, ils le savent très bien, il y a pas eu de brutalité. parce que les discussions ont eu lieu il y a pas eu de brutalité parce que le madame, la Première ministre a reçu combien de fois les syndicats. En quoi est-ce que le gouvernement aujourd'hui n'est-il pas autorisé ou fait pour faire ce débat, alors voilà. Ce texte, je le dis, il est d'abord nécessaire. Je crois que vous avez utilisé les rapports du COR qu'est ce que dit le corps le corps dit que dans la situation la plus favorable, il y aura 13 milliards de déficit en 2030 et qu'il faut les combler. Aujourd'hui vous dites que ce texte est injuste. Ce qui est juste demain c'est ce n'est pas de travailler plus aujourd'hui à juste ce qui est injuste et de laisser à nos enfants un système en perdition des retraites au rabais et une dette supérieure pour la France, voilà ce qui est injuste aujourd'hui voilà ce qui est un, alors je vous dis moi le chocolat. Je vous le dis franchement, maintenant. Nous allons voter ce texte parce que nous pensons qu'il était non seulement nécessaire mais qu'il est efficace aussi et ce que je vous le dis. Le ministre vous l'a redit l'autre jour ce texte une fois votée, vous pensez qu'il va laisser de la rancoeur de la fracture qui paiera aux élections. Moi quand je vote un texte ici je ne sais pas si ça va mais arranger électoralement ou pas électoralement. Ce que je sais et ce qu'il est bon pour des pays où est-ce qu'il est nécessaire et je le je le fais comme telle et demain je vous l'assure, Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre vous l'a dit, aucun gouvernement ne reviendra sur ce texte comme ça a été fait par le passé. Vous pouvez dire aujourd'hui ce que vous voulez-vous même si un jour vous accéder aux responsabilités parce que je ne souhaite pas, vous ne reviendrez pas dessus et vous aurez à redire les propos que vous avez tenu aujourd'hui. mes chers collègues ce président je vais conclure je voudrais à mon tour remercier ici remercier la Commission et les rapporteurs qui ont répondu avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'efficacité au fond aux arguments parfois a su que vous avez pu développer et remercier monsieur le Ministre ici qu'il a fait preuve d'une constance, d'une pédagogie d'une connaissance des dossiers que j'ai admiré moi même

Vous avez la parole. Si monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous y sommes. La droite sénatoriale s'apprête à voter cette réforme scélérate de recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Elle s'apprête à le faire main dans la main avec le gouvernement et les sénatrices et sénateurs de la majorité présidentielle. Vous avez pu parvenir à ce moment du vote malgré la contrainte de l'Arctique 47 1 de la Constitution. Parce que vous avez ensemble, gouvernement et majorité sénatoriale user de toutes toutes les procédures réglementaires et constitutionnel possibles et inimaginables pour accélérer les débats en censurant l'opposition de la gauche sénatoriale. Vous avez bloqué la démocratie. Le blocage c'est vous. Ce projet de loi est fondamental pour des millions de nos concitoyens et de nos concitoyennes ils veulent 2 années de retraite en bonne santé. Ah ces travailleuses et travailleurs qui, quel que soit leur corps de métier aspirent au repos. Ce projet de loi c'est aussi la nouvelle attaque compte les régimes spéciaux. Régimes pionnier qui concernent des professions rude voté la fin du régime spécial des électriciens et gaziers au moment où ils sont mobilisés dans des conditions très difficiles suite aux intempéries de ces dernières 48 heures est une insulte pour eux. Monsieur le Ministre, vous vous êtes empêtrés pour faire prendre des vessies pour des lanternes à votre peuple en affichant des avancées sur leurs carrières longues ou sur le revenu minimum de 1200 euros avancée qui s'avère lilliputiennes et même inconsistante. Vous avez multiplié dissimulation et contrevérités. Pour tenter de rendre acceptable. Votre texte, vous avez échoué. La toile de fond reste la même et personne n'est dupe. Vous voulez reculer l'âge de départ à la retraite. Ce projet de loi, vous l'avez aggravé mesdames et messieurs de la droite sénatoriale commande pas évoquer l'introduction par vos soins du ver dans le fruit des retraites avec votre amendement sur la capitalisation. Vous avez tomber le masque. Votre choix, c'est celui des fonds de pension. Vous vous attaquez au régime par répartition pour rendre de fait obligatoire le recours aux assurances privées. Nous l'avons dit d'entrée vous violer la Constitution à double titre, d'une part en empêchant le débat parlementaire et d'autre part, en mettant le principe républicain reconnus par le préambule de la Constitution 2946 issu du programme du Conseil national de la Résistance. Mais pour vous, Monsieur le Ministre. Il n'y a pas de principe. Votre priorité n'est pas leur bien-être c'est d'éviter de demander aux plus riches et au patronat. De payer de ne, de ne pas mettre la main à la poche parce que finalement il n'y a que ça qui vous intéresse. Avec vos nouveaux alliés de la droite sénatoriale. Vous avez refusé d'examiner sérieusement nos propositions d'Alter alternative au financement. Oui il est possible de. De rétablir la retraite à 60 ans véritable projet de justice sociale. À l'heure où des progrès scientifiques et technologiques. Partager les richesses partager le travail. Penser à un monde plus juste humain qui parle. Un projet de transformation sociale et écologique et qui n'alternative complète à votre projet libéral. Projet d'un vieux monde où seule la concurrence et le profit ne trouve grâce à vos yeux. Ce projet il grandit dans notre peuple que vous le vouliez ou pas. Il grandit en Europe et dans l'esprit de tous les peuples du monde. Cette réforme des des retraites. C'est une réforme rétrograde. Un projet de classe contre classe. Pour l'imposer. Vous avez donc choisi le coup de force anti-démocratique. Tous les moyens sont bons pour vous du détournement initial de la Constitution pour corseter le débat à l'application du vote bloqué au Sénat votre choix c'est l'autoritarisme. Emmanuel Macron refuse de recevoir les syndicats unis contre votre projet, affirme, dans une dérive bonapartiste assumer ne parler qu'au peuple. Mais enfin écoutez justement le peuple qui est vent debout. Vent debout qu'on va trop réformes écoutez-le une fois pour toutes le coup de force antidémocratique avec le non-vote de l'Assemblée nationale et le vote bloqué le vote. Du Sénat rend illégitime cette réforme des retraites rétrograde monsieur Macron veut s'adresser au peuple. Qu'il le fasse en organisant un référendum avec cette question êtes-vous pour ou contre le recul à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Pour ouvrir cette porte de sortie démocratique à la grave, très grave crise sociale et politique que nous vivons retirez votre projet retiré le avant que la colère populaire ne vous atteigne. Cette réforme et qui légitime. Je le redis, nous l'avons dit sans cesse sur les bancs de la gauche. Comme le brandissait une dame cet après-midi à la manifestation à Paris sur une pancarte. Je suis fatiguée. Laissez-moi laissez-nous enfin le temps d'être heureux et heureuses. Alors, retrait de cette réforme. À 64 ans et croyez-nous, croyez-moi, nous irons jusqu'au bout. bout. La parole est à notre collègue Henri Cabanel. Pour le groupe du Rassemblement démocratique. Et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci monsieur le président. Messieurs les. Les ministres, madame la présidente des affaires sociales, madame et monsieur le le rapporteur. Mes chers collègues. Mon groupe est déçu, déçu par cette mascarade de débat. Les yeux étaient rivés sur le Sénat. Nous aurions pu montrer la raison la conscience aux Français qui attendaient beaucoup de notre assemblée. Les Français qui, pour la sauvegarde du régime à répartition est essentielle. Après le spectacle désolant de l'Assemblée nationale. Nous aurions pu sortir ressortir grandit. Naïve My j'y croyais. Mais le scénario était écrit d'avance, les uns et les autres se rejetant la responsabilité de cet échec. Pourtant, pourtant il y a eu de moment rare trop rare de débats intéressants. Bien sûr, notre constitution, ainsi que notre règlement prévoit tous les cas de figure pour l'examen des textes de loi. Bien sûr, nous avons des droits pour des femmes dont Mais que dire des dizaines de prise de parole sur des rats, des rappels au règlement ou sur des dizaines d'amendements identiques bien avant l'article 17 sur l'âge de départ à la retraite. Ce n'est pas comme cela que l'on fait entendre nos voix ni qu'on gagne des voix. Bien sûr, le gouvernement n'a des droits aussi pour recourir aux 44 3 nous privant ainsi de débats dans la 2ème partie le Sénat aussi à travers son règlement, mais devait-on en arriver là. Que dire de la méthode, sur le véhicule législatif sur le rejet de la réforme par tous les partenaires sociaux. Ça j'oublier les nombreuses personnes dans les rues. Nous avions aussi des devoirs. Ceux de ne pas priver les Français d'un débat d'idées, de leur offrir la possibilité d'améliorer ce texte sur des sujets primordiaux. Je pense aux aménagements pour les carrières longues à l'amélioration des droits à pension pour les femmes, les étudiants, les sportifs, les personnes à situation d'handicap ou encore pour tous ceux qui s'engagent. À cet égard, j'espère que la main demain ne en groupe en faveur des pompiers volontaires résistera comme bout de beaucoup d'autres et que nous avons pu malgré tout faire adopter dans le brouillard de ces débats. Pour aller encore plus au fond de tout cela était-il trop demander de tout simplement débattre avec une envie véritable d'aller d'avancer, d'aller jusqu'au bout du texte. Notre devoir était de montrer notre sincérité. À mon avis, nous n'avons pas atteint ses objectifs, loin de là. L'image est désastreuse et notre responsabilité je pense et collégiale. Hé commun avec ceux-là réconcilier les Français avec la politique. Ils sont complètement écoeurés par ces méthodes est complètement déconnectée. On le serait à moins. Ces stratagèmes de vieilles politique ne serviront pas à notre comme à

Souvenons-nous tous des dernières élections. Ce qui s'est passé au Parlement sur ce texte laissera des traces. C'est bien dommage car je suis certaine qu'au fond. Tous ensemble nous sommes tous d'accord pour dire que notre démocratie Zyeux vaut mieux que cela. Au bout de ce tunnel de discussions. Chacun des membres de bon groupe votera cela hein. C'est selon ses convictions. Et je voudrais aussi remercier tous mes collègues qui pendant ces 10 jours ont été présents ainsi que remercier tous nos collaborateurs. Pour ma part je crois toujours à la nécessité d'une réforme. La stratégie d'évitement mise à oeuvre depuis 10 jours n'est pas à la hauteur des hein je. Reculer pour mieux sauter ne présage en rien de bon. Car c'est hypothéquer l'avenir dans notre système de retraite par 10 par répartition menacé par une logique démographique implacable. Un système auquel sont attachés nos concitoyens. Faut-il le rappeler, aussi, il est au coeur du pacte social de notre République. Il mérite d'être sauvé son équilibre ainsi que ses partenaires fondamentaux dont celui très important de la solidarité. Je vous remercie. Je vais donner la parole au président Claude Malhuret. Pour le groupe. Les indépendants. République et Territoires. Monsieur le président. Monsieur le président vous avez la parole. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur général monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues. En 1981 le premier président de gauche de la Ve République. A voulu faire croire aux Français que la situation de notre pays nous permettait d'abaisser l'âge de la retraite à 60 ans. Que nous serions des précurseurs et que les autres pays développés ne tarderaient pas à nous emboîter le pas. 10 ans plus tard après le déclassement économique des années 80. Et après que nos voisins européens et choisit le chemin exactement inverse qui consiste à augmenter l'âge de la retraite, parfois jusqu'à 67 ans. Un autre homme de gauche qui n'était pas lui un démagogue, Michel Rocard, expliqué qu'il fallait d'urgence revenir en arrière mais ajouté que ce retour à la réalité ferait chuter 4, gouvernement. Il n'était pas loin de la vérité. Depuis 30 ans. Plusieurs gouvernements ont tenté de réformer le système pour éviter les déficits abyssaux qui s'annonçait. Certains ont échoué, comme en 95. D'autres ont réussi au prix d'une part d'une impopularité certaines. D'autre part d'une limitation forcée de leurs objectifs qui n'ont jamais permis de résoudre le problème du déficit structurel due à la chute permanent du nombre de cotisants par rapport à celui des retraités.

Je suis d'ailleurs surpris. Que ceux qui ont défendu à l'époque cette réforme en constatant son inévitable impopularité et en sachant pertinemment qu'elle ne résoudrait les problèmes que pour un temps soit aujourd'hui dans le camp des adversaires acharnés de la réforme actuelle comme s'ils ignoraient sa nécessité. On dit souvent On dit souvent que l'on peut faire dire aux chiffres ce que l'on veut mais lorsque l'on parle d'un déficit dans le système de retraites de 150 milliards cumulés d'ici 10 ans comment nier la nécessité d'une nouvelle réforme. S'il est un objectif sur lequel nous pouvons tous nous mettre d'accord, c'est la préservation de notre régime par répartition et ce n'est pas en laissant croître le déficit que l'avenir de ce système sera assurée. Diminuer les pensions est inacceptable. Dans un contexte où l'inflation s'installe durablement et ronge le pouvoir d'achat. Augmenter les cotisations est inenvisageable dans un pays déjà médaille d'or au championnat du monde des prélèvements obligatoires. Reste donc le report de l'âge légal de la de départ à la retraite. C'est la solution retenue par ce projet de loi et c'est celle qui nous paraît la meilleure non pas la plus agréable ou la plus populaire mais la meilleure, en tout cas la plus juste et la moins mauvaise. Pendant de très longues heures nous avons entendu a de nauséabond. Plusieurs groupes de cette assemblée rabâcher d'autres pistes de financement. À un inventaire à la Prévert de taxes supplémentaires. Augmentation de la CSG, contribution exceptionnelle sur ceci ou cela. Taxe sur les robots et j'en passe et des meilleures. Mais au fond. Rien de cela ne devrait nous surprendre nous écoutons souvent ces mêmes propositions lors de l'examen du budget. Cette fois le prétexte et le financement du système de retraite. Mais l'objectif reste toujours le même taxer plus. Notre système de retraite, doit pouvoir s'équilibrait par les cotisations prélevées sur les salaires. Il a été construit ainsi il doit évoluer avec la réalité et non pas contre elle. Bien sûr, il est nécessaire de prendre en compte les situations particulières des Français ce débat au Parlement, été l'opportunité d'amender le texte en étant force de proposition. C'est pourquoi notre groupe apporter des amendements pour mieux protéger les plus précaires de nos concitoyens de tenir compte des carrières longues et de ceux qui ont commencé à travailler tôt, de ceux qui exerce un travail pénible tous les jours et qui doivent avoir le droit de partir plutôt en retrait des maires dont la carrière est parfois pénalisés par leur maternité, alors même que la natalité est un des facteurs clés de notre modèle par répartition des aidants qui vivent parfois des situations extrêmement difficiles et qui doivent être encouragées, ou encore des pompiers volontaires qui risquent leur vie et qui méritent notre reconnaissance malheureusement. Une partie du débat a été confisqué par la gauche. Sans avoir su convaincre nos concitoyens au cours des derniers scrutins. Sans avoir su proposer des solutions viables pour notre système de retraite. Elle n'a cherché qu'à retarder le débat. En déposant plus de 8000 amendements et sous-amendements en déposant des dizaines voire des centaines d'amendements de suppression sur chaque article. En déposant des amendements identiques qui déclinait un même dispositif en ne changeant qu'un seul chiffre en passant des heures entières de séance à faire des rappels au règlement qui n'en était pas vraiment les groupes de gauche ont choisi une stratégie d'obstruction délibérée et constante avec pour seul objectif la non d'adoption du texte. Il ne s'en sont d'ailleurs pas caché. Je suis navré de devoir le rappeler. Mais il n'y a pas en démocratie de minorité de blocage. Ce n'est pas parce qu'une minorité refuse de voter un texte qu'elle doit empêcher la majorité de le faire et je voudrais aussi rappeler que dans une démocratie. La loi ne se fait pas dans la rue mais au Parlement. Et au Parlement, la grande hypocrisie de ce débat, c'est que la gauche s'indigne aujourd'hui de l'utilisation de l'article 44 3 de notre loi fondamentale. Alors même qu'elle y a allègrement recouru pour faire adopter la réforme Touraine qu'elle portait en 2013 et 9 fois au cours du mandat de François Hollande. Nous n'ignorons pas que cette réforme est impopulaire. Et pour cause, elle exige des efforts supplémentaires de tous les Français, alors même qu'ils en fournissent déjà beaucoup. Mais c'est précisément parce qu'il s'agit d'une réforme aussi nécessaire que délicate. Que le Parlement se devait d'aller au bout de son examen. Ce n'est pas en fuyant nos responsabilités. Que nous ferons honneur à notre mandat et je voudrais après les orateurs qui m'ont précédé. Remercier notre président. Les ministres qui sont restés au banc pendant ces 10 jours. La présidente de la commission la rapporteure générale le rapporteur spécial et tous nos collègues dont la patience a été mise à rude épreuve et enfin l'ensemble du personnel du Sénat qui a participé à tous ses jours de discussions, l'avenir des Français est en jeu. Le texte que nous examinons depuis plusieurs jours est essentiel à bien des égards, car c'est la survie du régime par répartition qui est en cause parce qu'il s'agit d'un projet de loi nécessaire responsable et juste notre groupe votera en faveur de cette réforme.

Vous avez la parole. Si monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cette réforme des retraites est une des plus importantes de ce quinquennat quinquennat car à travers elle, c'est le système productif et le contrat social qui sont en jeu. C'est le travail, l'emploi, mais aussi les conditions de travail. C'est le temps libéré du travail subordonné la place des activités non marchandes. Ce sont toutes les problématiques sociales qui sont ici convoqués l'espérance de vie en bonne santé, le handicap, la part du travail dans la répartition des richesses. l'invalidité l'inaptitude c'est l'exclusion sociale, la précarité, la pauvreté qui ont été questionnés. C'est la place du prendre soin de l'autonomie des aidants. C'est la place des services publics et les conséquences de la baisse des effectifs et du gel du point d'indice des fonctionnaires, c'est la place des femmes des personnes immigrées et plus largement la question des discriminations sur le marché dans l'emploi qui sont mises en avant la retraite, ne peut être traitée avec une règle de 3 budgétaire. C'est un projet de société. Ces questions auraient mérité d'être débattue questionner, interroger, faire l'objet de controverse. Or nous nous sommes heurtés à un mur anti-démocratique pour bâillonner la minorité parlementaire. D'abord par le silence d'abord par le silence et la passivité de la droite sur nos propositions d'amendement pour résoudre le problème des ressources puisque le problème nous le rappelons ce n'est pas la dynamique des dépenses de retraites. Puis du 47 hein ou 44 3 de la Constitution du 40 de neuf de notre règlement. La mobilisation de tous les outils possibles pour imposer l'examen Express de nos amendements. Après le recours abusif aux irrecevabilité après le retrait d'amendements de la majorité de droite pour faire tomber les nôtres puis l'interdit d'expliquer nos votes dans un débat des dans un sénat dévitaliser de toutes les confrontations des arguments Ceci pour aboutir le plus vite possible au vote seul enjeu de la droite et du gouvernement. Un vote attends au plus vite la collusion de la droite sénatoriale et du gouvernement pour gagner une course de vitesse face à une mobilisation qui monte croissante inédite déterminé, une mobilisation d'une majorité de Français, de la quasi-totalité des actifs, des jeunes, des femmes de toutes les catégories socio-professionnelles et surtout de l'ensemble des syndicats de salariés, unis dans une intersyndicale historique et faisant du refus du recul de l'âge d'ouverture des droits de la retraite à la retraite. Une question non négociable. Une course de vitesse pour plier le débat car, jamais, jamais un texte n'a été autant impopulaire. La pièce qui s'est jouée au Sénat crée un précédent et dangereuse pour l'avenir de la démocratie parlementaire et pour la confiance de la population envers la démocratie représentative. Ce qui s'est produit ne profitera aucun de ces acteurs ni à la droite qui croit avoir enfin obtenu la victoire de leur projet régressif ni au gouvernement, qui se croit libéré d'une bataille alors qu'il a perdu tout soutien dans la population et donc toute légitimité sociale et morale. Toutes ces victoires arrachées par le pouvoir au corps défendant du Peuple sont rendues possibles par un glissement autoritaire qui nous éloigne des principes dont le corps politique se revendique pourtant la liberté et la démocratie. La façon dont le gouvernement impose son projet avec la complicité de la majorité conservatrice du Sénat annonce une aire libérale où l'extrême droite ne saura que la seule bénéficiaire car nous le savons. Cette réforme antisociale des retraites n'était pas nécessaire. Et le déficit. Il a été construit par la non volonté d'y allouer des ressources. L'ensemble de nos propositions ont été balayés alors qu'elles étaient juste socialement et durable, tant sur le plan financier qu'environnemental, des 18 milliards ne seront générés que par le monde du travail nullement sur le capital nullement sur les très hauts patrimoines nullement sur les bénéficiaires depuis de 2017 du désarmement fiscal. Uniquement sur les travailleurs. Travailleuses et des travailleurs qui verront s'éloigner l'horizon de leur vie hors travail. Ces années de travail supplémentaires ne sont plus permises par l'augmentation de l'espérance de vie. Elles sont prises sur la durée de la retraite qui diminue désormais. On se sera alors le travail plus proche de la mort. C'est ce qui fonde inconsciemment la force du refus. Ces années de plus sont prix sur l'espérance de vie en bonne santé ou prolonge une situation de pauvreté, de précarité. Pour faire passer cela. Nous avons assisté à une exaltation du travail comme si tout travail était pas construction par définition émancipateur et comme s'il refusait de le prolonger sans fin était la négation de sa place. Venant d'un gouvernement qui nient la pénibilité du travail. Rien de nouveau. À défaut de changer les choses ont changé, les mots pour les maçons, les aides à domicile, les chauffeurs de bus, les égoutiers, les professeurs, les soignants, les agriculteurs, les employés et les ouvriers le travail et surtout à partir d'un certain âge peut être si une offre une souffrance qui abîme les corps et les esprits et toutes les statistiques montrent que cela est de plus en plus vrai. Or, qu'avons-nous pour elle et eux dans ce texte, à part un index non contraignant que le Conseil du constitutionnel risque d'exclure comme cavalier social. Quant aux mesures d'atténuation de la brutalité de cette réforme. Elles ont été évoquées dans un combat sans contradictoire et c'était mieux vu des mensonges. Quant aux 3 milliards annoncés pour l'incapacité. Permanente, c'est un mensonge. Il n'existe pas puisque rien ne change sur ce point vous voter cette réforme contre le peuple vous voter cette réforme au nom de l'avenir avec un logiciel du passé. Le sens de l'histoire c'était et cela reste la retraite à 60 ans, c'est la baisse du temps de travail et la transformation de notre modèle de production et de consommation, c'est la reconnaissance des activités selon leur utilité sociale et non au profit de l'accroissement ça sans fin de richesse de quelques ça ne voteront pas cette réforme, pas uniquement pour les raisons que nous avons développé mais parce que nous avons un autre projet, celui de l'écologie sociale ce soir la bataille au Sénat aboutit à un vote de la droite pour sauver le gouvernement mais la bataille contre c'est tout continue et autant qu'il le faudra. La gauche et les écologistes la mèneront jusqu'au retrait.

monsieur le président. Cette réforme a été présentée comme la mère de toutes les réformes et vous savez que, pour nous en tout cas elle constituera une. Une régression sociale pour plusieurs millions de nos concitoyens qui seront malheureusement à payer un impôt mais un impôt sur leur vie de de retraite. C'est une forme donc essentiel. Mes chers collègues. Et nous pensons au nom des 3 groupes de gauche ici présents et mes collègues. Et Gontard et tous les collègues ici présents 30 signataires demandent l'application de l'article 51 de notre règlement. À savoir que la présence dans l'enceinte du palais de la majorité absolue des sénateurs est nécessaire pour la validité des votes sauf en matière de fixation de l'lors du jour donc. Monsieur le Président, je sollicite de votre part cette conversation cette constatation éventuelle. Bien monsieur le président. le président. S'il vous plaît. Je suis saisi d'une demande écrite. Monsieur le Président. Par vous-même de vérification du quorum. En application de l'article 51 alinéa 3 du règlement. La constatation du nombre des prisons est effectuée sur la demande écrite de 30 sénateurs, dont la présence doit être constatée par appel nominal. Il doit donc être procédé à l'appel nominal des signataires de la demande de vérification du quorum et les huissiers vont donc effectuer cet appel à vous.

Cieux Yan Chantrel. Monsieur Rémy Cardon. Madame Laurence Cohen. Monsieur Thomas Dossus. Monsieur Jérôme Durain. Monsieur Jacques Fernique. Madame Corinne Ferré.

Madame Marie-Pierre Monnier. Monsieur Franck Montaugé. Madame Raymonde Poncet Monge. Madame Émilienne Pumerole. Monsieur Lucien Stones, Jon. Monsieur hein. Rachid Temal. Monsieur Jean-Claude Tissot. Madame Sabine von. Madame Mélanie Vogel. Mes chers collègues, je constate. La paella. Je constate. Que la présence d'au moins 30 sénateurs. Est effective. Il peut être procédé à la vérification du quorum. Je vais procéder à la vérification du quorum j'invite donc en application de l'article 51 alinéa de du règlement. De secrétaire à venir m'assister en l'occurrence monsieur Jacques Grosperrin et monsieur Jean-Claude Tissot.

Monsieur le Président Kader. Pouvez-vous venir à mes côtés avant que je procède.

Je vais donc mettre au revoir. S'il vous plaît. Je vais mettre aux voix les Arctic 9 à 20, modifié par les amendements adoptés le Sénat. À l'article 9. Et ceux proposés ou acceptés par le gouvernement ainsi que l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023. Le. Je rappelle qu'en application de l'article 59 du règlement le scrutin public et de droit. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos.

Monsieur le Ministre, dans deux secondes. Mes chers collègues. Nous sommes parvenus. Au terme de ce débat très dense. Dans lequel. Chacun s'est exprimé. Depuis le jeudi 2 mars. Nous avons siégé. 10 jours. Bonsoir. Et quasiment autant de nuit en continu. Pour un total de plus de 100 heures de débats. Nous avons enregistré un nombre record d'amendements de sous-amendements, 8900 au total. Le débat a eu lieu à débat qui ait pu être éclairés où chacun a pu affirmer sa position sur chaque parti, chaque apport du. Sur l'article 7. Qu'on peut qualifier de coeur du réacteur dont nous avons engagé la discussion le mardi 7 mars ou soit. Nous avons eu 63, prise de parole sur l'article avant la présentation des 77 amendements de suppression d'articles. Nous avons débattu. Plus de 13h sur ce seul article 7. Les règles de procédure et celles fixées par la Constitution. Nous conduisent à achever l'examen de ce texte dans le délai de 15 jours imparti au Sénat. Par delà nos divergences. Qui sont profondes. Je crois que nous avons pu mettre l'empreinte du Sénat sur ce texte. Je voudrais saluer le travail approfondi. De madame la rapporteure générale et du rapport. Auteur de la branche vieillesse et de la présidente de la commission. Des affaires sociales. Parce Parce que eux ils ont fait les chanteurs. Plus le travail en commission, plus de travail préparatoire. Je voudrais saluer. Le travail de l'ensemble des membres de votre commission, madame la présidente de la commission, ainsi que celui des collègues sénateurs de l'ensemble des groupes. Je voudrais vous remercier, monsieur le Ministre pour messieurs les Ministres pour. Votre présence tout au long de nos débats, ainsi que pour la pédagogie. Vous avez. Démontré au cours de de ce débat. Ce travail va maintenant se poursuive son chemin. En commission mixte paritaire. Avant de nous revenir la semaine prochaine. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remercions. Mes chers collègues permettez-moi de remercier particulièrement. Les vice-, président du Sénat qui ont été à la tâche et qui se sont répartis dans leur diversité diversité. C'est plus de 100 heures de débats. Moi aussi je voudrais. Associer l'ensemble. J'allais dire particulièrement du service législatif du service de la commission des affaires sociales qui ont été vraiment dans une tâche. Exceptionnel. Pour certains c'était leur baptême du feu. Pour d'autres l'apogée presque d'un. Première étape de carrière en vous souhaitant le meilleur chère madame. Pour la suite. En tous les cas je voulais vous dire que j'ai le sentiment d'être le président d'une institution qui a joué son rôle et qu'il a joué avec engagement responsabilité avec pour seule ligne de crête, quelles que soient nos sentiments l'intérêt du pays et l'intérêt des Français. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président. Merci pour vos mots mesdames et messieurs les sénateurs, madame la présidente de la Commission. Mesdames et Messieurs, Mesdames, trois mots à mon tour d'abord pour vous dire qu'. Avec mon collègue Franck Riester avec Gabriel Attal, qui était présent à nos côtés pour les Arctic financier. Je voudrais adresser tous mes remerciements à madame la présidente et mesdames et monsieur le rapporteur pour la qualité des des relations que nous avons entretenu pour les travaux préparatoires. Les échanges ont parfois été vifs sur porteur. Parce que nous n'avons nous avions quelques divergences et il en reste sur ce texte. Mais je crois que nous avons fait cela dans un climat constructif dans un climat de travail et avec la volonté. De porter un texte de faire en sorte que chacun puisse se retrouver et espérer qu'à la fin de tout ce processus, le texte soit. Adopté et qu'il puisse être le meilleur possible. Je voudrais remercier tous les sénateurs tous les sénateurs qui ont participé à ce débat des présidents de groupe et les sénateurs. Parce que je pense que chaque contribution a été utile et que les groupes ont pu faire valoir des positions. Les sénateurs ont pu faire valoir des positions et à travers ses positions à travers les amendements qui ont été adoptés. Le texte a pu être enrichi sur la question des orphelins sur la question des mères de famille sur la question des agriculteurs des sapeurs-pompiers du rachat de trimestres encore des élus locaux. Je sais combien madame la rapporteure pour avis est particulièrement attaché. Nous avons enrichi ce texte et nous devons, je crois, espérer que la suite du débat parlementaire, la commission mixte paritaire les étapes qui suivront, permettre de l'enrichir encore pour que ce texte puisse ainsi poursuit son son chemin législatif. La, la 2ème, chose que je voulais vous dire à vous tous et peut être à vous encore plus particulièrement Monsieur. Monsieur le Président, c'est que beaucoup d'entre vous. On peut être pris un peu l'habitude de me voir, depuis quelques années au travers des différentes fonctions que j'ai exercé et beaucoup d'entre vous savez que le savent que j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver le sénat débattre au Sénat et que j'apprécie à la fois la, la qualité de vos travaux mais aussi leur calme et comme. Les sentiments comme le plaisir. Le plaisir intellectuel la satisfaction intellectuelle ce sont des sentiments relatif qui se mesure toujours à l'aune du déplaisir que l'on peut connaître par ailleurs j'ai encore plus apprécié cette fois-ci. Et enfin, Monsieur le Président, permettez-moi de, de m'associer à à vos mots pour. L'ensemble des services du Sénat. Ce n'est peut-être pas la coutume, mais je voudrais à la fois saluer la qualité l'intensité du travail mais aussi remercier l'ensemble des services du Sénat l'ensemble des agents pour la très grande gentillesse avec laquelle ils accueillent les membres du gouvernement. Nos équipes combien ils peuvent aussi en même temps qui vous accompagne dans leurs fonctions. Nous faciliter le travail ici remercier l'ensemble des équipes qui m'accompagnent sur ce texte. Évidemment les les services du ministère du Travail. Les services du gouvernement mais vous comprendrez que j'ai une attention toute particulière pour mon cabinet. Ils ont un engagement et un investissement que dont je suis le témoin le plus privilégié et qui est absolument absolument remarquables. Et enfin dernier point pour vous dire que. Je suis particulièrement heureux parce que parlementaire depuis 2017 quand le Parlement vote et quand le, quand le Parlement légifère. Merci à tous. Merci, monsieur le Ministre. Merci messieurs les ministres. de participer à l'exercice de compétence de l'État. La séance est levée.